mes chers collègues, alors que l'armée russe intensifie, en ce moment même, ses attaques en bombardant Kharkiv, en resserrant son étau autour de Kiev, en donnant l'assaut à Marioupol et en prenant pour cibles les populations civiles, je souhaiterais que nous rendions, ensemble, hommage à la résistance du président Zelensky, des autorités et du peuple ukrainiens, qui affrontent avec bravoure l'invasion de leur pays.

C'est pour cette raison que j'ai voulu la présence, dans notre hémicycle, du drapeau de l'Ukraine, aux côtés des drapeaux français et de l'Union européenne. Je voudrais adresser, en votre nom à tous, un salut fraternel au président de la Rada de la République d'Ukraine, M. Ruslan Stefanchuk, et aux collègues parlementaires ukrainiens. Le parlement ukrainien a toute sa place dans la grande famille du parlementarisme européen. J'aurais dû m'entretenir cet après-midi même par téléphone avec le président de la Rada,

des parlements des vingt-sept États membres de l'Union européenne et du Parlement européen ont adopté, par consensus, une déclaration solennelle de solidarité à l'égard de l'Ukraine. Cette déclaration intervenait dans le cadre du volet parlementaire de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Mais au-delà de la manifestation de solidarité, la déclaration adoptée s'est voulue exigeante. Elle a demandé aux gouvernements européens et à la Commission européenne d'intensifier encore les mesures prises à l'encontre de la Russie et d'amplifier le plan de soutien au Gouvernement ukrainien, qu'il s'agisse de l'aide humanitaire, des mécanismes de protection civile ou de la fourniture à l'Ukraine de tous les moyens nécessaires, y compris militaires. En En cet instant de gravité, il importe d'être à la hauteur des circonstances, car les destins de l'Ukraine et de l'Union européenne sont intimement liés : en Ukraine se jouent aussi la sécurité et les valeurs de l'Union européenne.

en décidant, dans la nuit du 23 au 24 février, de déclencher une attaque militaire massive contre l'Ukraine, la Fédération de Russie a commis un acte de guerre qui enfreint toutes les règles du droit international, rompt avec tous ses engagements et bafoue les valeurs de paix et de liberté sur lesquelles le continent européen a construit son équilibre depuis plusieurs décennies. Comme le Président de la République l'a souligné, nous faisons face à une situation de guerre, mais également à un tournant dans l'histoire de l'Europe et de notre pays. Je veux le redire ici d'emblée : la France condamne de la manière la plus absolue cette agression cynique et préméditée. En ces instants tragiques, je veux redire tout notre soutien au peuple ukrainien qui vit des moments terribles, ainsi qu'à toutes les victimes de ce drame, absolument inconcevable entre deux pays voisins en Europe au XXI siècle. Je veux également dire mon admiration au président Zelensky qui, depuis Kiev assiégée, mène le combat et fait face avec courage, responsabilité et dignité.

Cette équipe, sous l'autorité de notre ambassadeur, Étienne de Poncins, oeuvre dans des conditions particulièrement difficiles. Pour des raisons de sécurité, elle s'est

aux présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale et aux présidents de groupe et des commissions compétentes des deux assemblées de réunir sans délai un comité de liaison qui nous a permis de partager, vendredi dernier, des informations importantes et de répondre à l'essentiel des questions qu'ils ont bien voulu nous soumettre. J'ai invité hier, dans le même esprit, les candidats à l'élection présidentielle. J'ai également souhaité répondre à la demande légitime que la représentation nationale tout entière puisse s'exprimer sur ce sujet de la plus haute importance,

Mesdames, messieurs les sénateurs, la France n'a pas ménagé ses efforts ces dernières semaines et ces derniers mois pour faire valoir, jusqu'au bout, la voie de la raison et de la paix. Ce faisant,

en 2013, et ensuite avec les accords de Minsk de 2014, signés alors que le président Hollande était à l'Élysée. En tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, en tant que présidente en exercice du Conseil de l'Union européenne, au regard aussi de ce que sont ses valeurs et l'idée qu'elle se fait de la paix et du mode de résolution des conflits, la France se devait, se doit, d'assumer son rôle. Les initiatives prises par le chef de l'État se sont multipliées, en liaison étroite avec nos partenaires européens et les États-Unis. Ces efforts n'ont pas abouti. Vladimir Poutine a non seulement déchiré les accords de Minsk, mais il a aussi rompu tous les engagements qu'il avait pris dans les derniers jours.

Nous observions avec nos partenaires et alliés le déploiement progressif d'un dispositif militaire massif en Biélorussie, aux frontières de l'Ukraine, en mer Noire : plus de 150 000 hommes, équipés des moyens les plus modernes. Ce dispositif militaire, le président russe nous assurait qu'il se retirerait une fois les exercices terminés, tout en appelant au dialogue diplomatique sur des garanties de sécurité pour la Russie, et tout en répétant que la Russie ne s'apprêtait pas à envahir à envahir l'Ukraine. Vladimir Poutine a menti. Il a menti à la communauté internationale, il a menti au Président de la République, il a menti à son propre peuple. Non, aucun génocide n'a eu lieu contre les populations russophones du Donbass. Non, il n'y a pas d'armes nucléaires sur le sol ukrainien. Non, M. Zelensky n'est pas à la tête d'un régime nazi, terme particulièrement infâme quand il est appliqué à un pays pleinement démocratique. La suite, vous la connaissez : le 21 février, les masques sont tombés. La reconnaissance par le président de la Fédération de Russie des deux régions séparatistes de l'est de l'Ukraine, l'ordre donné aux forces russes d'occuper ces territoires et l'invasion de l'ensemble du territoire ukrainien depuis la Russie, la Crimée et la Biélorussie constituent le premier acte de cette crise qui sera sans doute longue. Vladimir Poutine a ainsi fait le choix de la guerre. Il a fait le choix de vouloir inverser le cours de l'Histoire et de revenir sur les acquis qui avaient suivi la fin de l'Union soviétique. Il a pris le prétexte de la situation dans la région du Donbass pour violer la souveraineté territoriale et chercher à renverser le gouvernement légitime d'un pays de 44 millions d'habitants. Face à cette agression inacceptable, il convient de réagir dans l'unité et dans la durée pour, à la fois, soutenir nos amis ukrainiens et ne pas laisser cet acte de guerre sans réponse ni conséquence.

fermeté. D'abord, par respect pour le droit international, dans l'enceinte des Nations unies : la résolution présentée en urgence devant le Conseil de sécurité n'a pas été adoptée en raison du veto russe, mais elle a permis de démontrer l'isolement de la Russie, de même que les échanges, très intéressants, qui ont suivi en Assemblée générale et qui ont donné lieu à une condamnation extrêmement large et ferme par la communauté internationale. Ensuite, par la mise en place de plusieurs trains de sanctions que nous avons voulu prendre très rapidement. Le Conseil européen, sous présidence française, a ainsi approuvé trois paquets de sanctions les 23, 25 et 27 février. Ces mesures prises en coordination avec nos alliés couvrent un éventail large des activités économiques russes. Tout d'abord, nous avons décidé d'assécher la capacité de financement extérieur de l'économie russe. Depuis hier, quatre heures du matin, toutes les transactions avec les réserves de la banque centrale russe sont interdites et ses avoirs détenus à l'étranger sont gelés. Cette mesure est complétée par l'interdiction imposée à la majorité des banques russes d'accéder à la messagerie de transmission des paiements Swift. Ce paquet de sanctions financières est inédit par son ampleur et ses effets sont déjà palpables : le rouble a dévissé de près de 30 % à l'ouverture des marchés lundi matin. L'Union européenne a également fermé l'intégralité de son espace aérien aux aéronefs et aux compagnies aériennes russes, y compris l'aviation d'affaires. En outre, les avoirs et les ressources économiques détenus et contrôlés par les personnes sur lesquelles s'appuie le pouvoir de Vladimir Poutine ont été gelés.

Vladimir Poutine fait d'ailleurs partie de la liste des personnes sous sanction, tout comme Sergueï Lavrov. les différentes coopérations entre l'Union européenne et la Russie dans les domaines industriel, scientifique, culturel ou sportif sont suspendues.

Les échanges se poursuivent pour aller plus loin. Nous y sommes prêts. L'essentiel était d'agir rapidement, de bien cibler nos mesures pour qu'elles produisent un effet massif sur l'économie russe, à court terme bien sûr, mais aussi et surtout dans la durée, quitte à les durcir encore au cours des prochains jours. Évidemment, ces sanctions ne seront pas indolores pour les économies européennes. Nous le savons et nous vous proposons de l'assumer, sauf à se contenter de mesures sans réelle portée. Bien sûr, nous savons que la Russie arrêtera à son tour des contre-mesures

Le bouclier tarifaire sur les prix de l'énergie a ainsi permis de consacrer plus de 16 milliards d'euros à la protection de nos concitoyens et de nos entreprises face à la hausse des prix de l'énergie.

Mais c'est bien la Russie qui va souffrir le plus des conséquences de ces sanctions. La guerre unilatérale et injustifiée que Vladimir Poutine a déclenchée doit avoir un coût élevé pour lui et ses soutiens. Le deuxième principe de notre action, c'est la solidarité avec le peuple, le gouvernement et le parlement ukrainiens. Cette solidarité, le Président de la République l'a réitérée au président Zelensky lors de leurs entretiens quasi quotidiens.

dans ce cadre, 33 tonnes de matériel humanitaire parties de Paris sont déjà arrivées à la frontière ukrainienne. Les acheminements se poursuivent cette semaine, incluant de l'aide médicale La France soutiendra aussi les pays frontaliers de l'Ukraine qui accueilleront les réfugiés et nous proposerons, dans le cadre de la présidence du Conseil de l'Union européenne, qu'un dispositif de solidarité permette une juste répartition répartition des efforts d'accueil de ces réfugiés entre les pays de l'Union. Bien entendu, nous y contribuerons nous-mêmes. Je veux aussi souligner la forte mobilisation spontanée de nos concitoyens,

Troisième principe de notre action, l'unité. Tout ce que nous faisons- c'est une condition d'efficacité -, nous le décidons conjointement avec nos partenaires au sein de l'Alliance atlantique comme de l'Union européenne.

Cette unité, cette rapidité, cette intensité ont surpris, y compris, sans doute, le président Poutine. Cette unité, cette rapidité, cette intensité sont inédites. Nous pouvons collectivement en être fiers.

au coeur du prochain Conseil européen des 10 et 11 mars prochains qui examinera notamment le projet de boussole stratégique que nous avions,

c'est le maintien du dialogue. Comme je vous l'ai déjà dit, la diplomatie française n'a jamais ménagé ses efforts pour éviter cette crise et chercher inlassablement le chemin de la désescalade. Le Président de la République s'est personnellement engagé et continue de le faire. Nous restons persuadés que la diplomatie a encore toute sa place pour mettre fin à la guerre et nous continuerons de dialoguer avec tous les protagonistes de cette crise, sans relâcher nos efforts et sans céder sur les principes du droit et du respect de la souveraineté des États. Ce dialogue est indispensable, mais si Vladimir Poutine ou ses collaborateurs souhaitent négocier, ils doivent d'abord faire taire les armes. Encore hier, le chef de l'État s'est entretenu longuement avec le président russe. Il a réitéré la demande de la communauté internationale d'un cessez-le-feu immédiat. Il a appelé au respect du droit international humanitaire et de la protection des populations civiles comme de l'acheminement de l'aide, conformément à la résolution portée par la France au Conseil de sécurité des Nations unies. Mesdames, messieurs les sénateurs, cette crise sera longue et aura des conséquences majeures sur l'avenir de l'Europe, mais pour autant c'est bien le droit, la paix et la démocratie qui devront à la fin en sortir vainqueurs. Nous assistons au premier acte. Il n'est pas terminé et, sans surprise, il fait apparaître le déséquilibre des forces en présence, mais aussi mais aussi le courage admirable du peuple ukrainien et la mobilisation inédite de la communauté internationale. Nous avons toujours été clairs et nos amis ukrainiens l'ont d'emblée compris : un pays comme la France ne peut recourir à la force que si elle est directement attaquée ou dans le cadre des systèmes d'alliance dont elle fait partie. L'Alliance atlantique dont nous sommes membres est une alliance défensive. Elle se défend lorsque l'un de ses membres est agressé, et l'Ukraine n'est pas membre de Mais il n'y a aucun doute sur le fait que nous serions amenés à nous engager militairement pour la protection de nos alliés de l'Europe de l'Est si le conflit devait connaître d'autres extensions au-delà du territoire ukrainien, dans les pays membres de l'Alliance. Le Président de la République a d'ores et déjà décidé de renforcer notre participation au dispositif de l'OTAN dans les pays baltes, en Pologne et en Roumanie. Tout en restant engagée dans l'approfondissement de l'Europe de la défense, la France tient sa place de membre actif, solidaire et impliqué dans l'Alliance atlantique. je rappelle que nos forces armées participent sans interruption depuis plusieurs années à la réassurance de nos alliés orientaux, notamment dans les pays baltes où notre engagement va se poursuivre

ici rappeler à la représentation nationale et à l'ensemble de nos concitoyens que, si nous le pouvons, c'est parce que le Président de la République a su donner depuis 2019 une inflexion forte aux moyens affectés à notre défense nationale.

tout mettre en oeuvre, collectivement, pour écrire les actes suivants de cette crise. Elle va s'inscrire dans le temps long.

abreuvé par une propagande médiatique qui travestit la réalité des faits. Je ne suis pas certain que ce soit le destin qu'il ait choisi, car le peuple russe est un grand peuple. Les efforts de guerre qu'il faudra payer, les sanctions économiques subies, la mise au ban des nations vont appauvrir et isoler la Russie au détriment de son peuple qui n'a évidemment pas été consulté par son président. Nous devons nous adresser au grand peuple russe et clairement mener la bataille de la communication, dans un cadre partenarial, comme nous avons commencé à le faire avec les chaînes d'information, ou plutôt de désinformation, contrôlées par le pouvoir russe. Mesdames, messieurs les sénateurs, vous l'aurez compris, l'agression de l'Ukraine par les forces de Vladimir Poutine va bien au-delà d'un simple conflit entre deux pays. Cette agression, qu'il qualifie dans son narratif d'« opération militaire », est en réalité une atteinte majeure aux principes les plus fondamentaux du droit international, de la souveraineté et de l'intégrité des États. Ces bruits de botte à l'est de l'Europe nous replongent dans des périodes de l'histoire que nous pensions durablement derrière nous. À cela, nous voulons répondre différemment et collectivement, en privilégiant la plus grande fermeté dans nos actions, l'unité avec nos alliés et nos partenaires européens et surtout la solidarité sans faille avec le peuple ukrainien et ses dirigeants, qui, par leur résistance, leur dignité, leur courage, forcent notre admiration et nous obligent. Nous devons être à leurs côtés pour les soutenir, aujourd'hui et demain, par tous les moyens utiles. À la fin des fins, nous devrons toujours chercher à privilégier l'arme de la diplomatie, la seule qui vaille dans nos démocraties. Nous le ferons, en nous adressant aux peuples russe et ukrainien, deux peuples matures auxquels nous rappellerons incessamment que la voie de la force et de l'impérialisme finit toujours par conduire à l'impasse. Si aujourd'hui les chars russes envahissent Kiev et non pas Budapest ou Prague, c'est justement parce que l'Europe a su construire avec ses partenaires, autour d'aspirations communes, un ensemble sûr, uni, prospère. Le peuple ukrainien aspire, dans sa majorité, à rejoindre cet ensemble, à s'associer à ce mouvement. Ce mouvement reprendra assurément, car c'est le sens de l'Histoire. Acte

Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, madame la ministre, messieurs les ministres, mes chers collègues, collègues, la guerre est de retour en Europe et, avec elle, ces images que nous pensions appartenir définitivement au passé : les sirènes hurlantes dans les villes ukrainiennes, la population qui se masse sous terre et les civils- femmes, enfants, vieillards -qui sont jetés sur les routes de l'exode.

sur l'initiative du chef de l'État, monsieur le Premier ministre. En renforçant les positions orientales de l'OTAN en Pologne, en Estonie, mais aussi en Roumanie, nous envoyons à la fois un message de détermination et de fermeté, mais surtout un message d'unité. J'observe au passage que le président de la Fédération de Russie aura finalement réussi

la France n'était elle-même que lorsqu'elle portait une part de l'espérance du monde. Aujourd'hui, la France porte une part de l'espérance du monde, ou plutôt une part de l'espérance ukrainienne. mes chers collègues, nous sommes tous ukrainiens. Vive la République, vive la France, et surtout vive l'Ukraine libre !

Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, madame la ministre, messieurs les ministres, mes chers collègues, le 24 février, la Fédération de Russie a décidé, sur l'ordre de son président, Vladimir Poutine, l'invasion d'un autre pays souverain, l'Ukraine, en violation flagrante du droit international. Une guerre se déroule sous les yeux du monde. Poutine a mis tout en oeuvre pour cacher ses intentions, et désormais les morts et les blessés. Mais le courage des Ukrainiens, notamment celui du président Zelensky, permet à la communauté internationale

Nous pensons également à la communauté française résidant en Ukraine. Comment ne pas y penser, nous qui pour beaucoup sommes liés par nos récits de vie à cette Europe de l'Est si souvent malmenée à travers l'histoire ?

Toutes ont un jour trouvé un foyer dans notre pays. Alors, en m'exprimant à la tribune de la Haute Assemblée de la République, mes pensées sont imprégnées d'une émotion singulière. Nous mesurons en ces instants que la guerre n'est pas le prolongement naturel de la politique, mais bel et bien la somme de la déraison et de la haine.

L'automne 1956 et le printemps 1968 avaient vu les cortèges d'espoirs décimés sous le poids des blindés et des bottes. Nous ne pouvons pas rester spectateurs de la répétition de l'Histoire et de ses pages le plus sombres.

Nous mesurons le poids de ses mots et notre engagement républicain doit être total au service de la construction de l'Europe. Ces derniers temps, jusque dans notre propre pays, nous constatons la tentation d'opposer les Français entre eux, ou d'attiser les communautés entre elles. Nous combattrons cela avec la même énergie elles. Nous combattrons cela avec la même énergie ! Le patriotisme ne se mesure pas aux harangues et aux coups de menton. Ceux qui crient à une prétendue identité surannée sont aux abonnés absents quand il s'agit de tenir le drapeau. En cela, ils ne sont que les héritiers de ce que la France a produit de pire à travers son histoire. produit de pire à travers son histoire. Lorsque l'on se revendique français, enfant du pays des Lumières, il n'y a pas de place possible pour une parole politique dont le projet est justement la destruction méthodique de la liberté. Je le dis clairement

ceux d'une Europe en guerre permanente et ceux d'un continent qui prenait les armes tous les trente ans. Nous le réaffirmons ici : le projet de renaissance des anciens empires sur la scène internationale est l'une des sources les plus inquiétantes pour la stabilité du monde et pour la paix. La mémoire de deux guerres mondiales a conduit l'humanité à se doter d'organisations internationales, afin d'éviter que les attitudes expansionnistes et paranoïaques de quelques dirigeants ne débouchent sur de tels drames. Poutine omet

Mais il n'y a pas de fatalité. Le meilleur de la Russie se trouve dans le coeur du peuple russe. Je veux saluer le courage de ces femmes et de ces hommes

Je salue également les mouvements sportifs et culturels, qui ont su prendre leurs responsabilités. Nous disons au peuple russe, trop souvent manipulé, que la France, l'Union européenne et le monde se tiendront à leurs côtés pour reconstruire la paix le moment venu. Oui, nous voulons la paix, la tempérance, la sérénité pour notre génération et les générations futures, ici et partout dans le monde ! Les opinions publiques nous y invitent. C'est grâce au soutien des opinions publiques que l'Union européenne progresse comme elle ne l'avait pas fait depuis si longtemps. Nous savons aujourd'hui, à l'épreuve des faits, que l'Europe de la défense ne doit plus être un voeu pieux. Sans porter atteinte à la souveraineté des États membres, elle est la garantie d'une véritable diplomatie européenne. Elle en représente la crédibilité et l'indépendance.

D'ores et déjà, je propose que nous accueillions les réfugiés ukrainiens dans les meilleures conditions possible en leur octroyant provisoirement les mêmes droits que ceux détenus par les citoyens européens, afin qu'ils puissent se reconstruire un futur.

Je pense à ces femmes, à ces enfants et à ces personnes âgées, et je dénonce l'ignominie des propos tenus hier matin par l'un des candidats d'extrême droite à l'élection présidentielle française.

Certains en discutent l'efficacité réelle ; pour notre part, nous considérons qu'elles sont nécessaires. Nous demandons également au Gouvernement de prendre l'engagement ici de ne pas reconnaître, s'il devait advenir, un pouvoir fantoche en Ukraine, marionnette de la Russie. Ces sanctions sont nécessaires, même si elles demanderont des efforts en retour. Nous devons les anticiper dès aujourd'hui : toutes les inégalités sociales, qui sont déjà insupportables, pourraient s'accentuer si l'on ne s'y attaque pas avec détermination. Pour compenser les conséquences économiques à venir des décisions que nous avons portées, il faut nous atteler dès maintenant à construire un bouclier de justice sociale qui protégera les Français, particulièrement les plus fragiles, éventuellement en demandant un effort exceptionnel aux ménages qui ont le plus profité de ce quinquennat. Cette question sociale n'est pas que conjoncturelle, mes chers collègues. Il faut avoir conscience que les inégalités sont le creuset des crises à venir, comme le sont aussi les questions environnementales et énergétiques. Nous devons prendre dès aujourd'hui la mesure des défis qui sont devant nous

nous recherchons le retour à la paix. Les pays baltes, les Balkans et l'ensemble des pays à proximité géographique de la Russie doivent savoir que nous sommes à leurs côtés. Cet engagement pour la paix va de pair avec la confiance dans nos armées. Mon groupe a toujours soutenu le renforcement de nos capacités afin qu'elles aient les moyens opérationnels de mener toutes leurs missions de protection. Vous pouvez compter sur nous, monsieur le Premier ministre, pour continuer dans cette voie. Je salue d'ores et déjà l'engagement de nos militaires, prêts à toute éventualité, et je leur exprime notre profond respect.Car tout démontre que c'est dans le rapport de force, y compris militaire, avec Poutine que la voie de la diplomatie pourra être retrouvée. Lui seul nous oblige à réagir ainsi. Ses crimes contre les civils en Ukraine relèveront aussi, un jour, de la Cour pénale internationale : je demande que la France prenne toute initiative en l'espèce. Aucun traité ne saurait être arraché par la force ; c'est d'égal à égal, sous la protection de l'ensemble de la communauté internationale rassemblée au sein de l'Organisation des Nations unies (ONU), que l'Ukraine et la Fédération de Russie doivent définir les modalités de leur coexistence. Je souhaite aussi attirer l'attention sur la nécessité du respect du Parlement, monsieur le Premier ministre. Nous sommes une démocratie- c'est aussi notre différence -, et l'exécutif a un devoir d'information du Parlement en cette période de crise sur la question des moyens à apporter à l'Ukraine, tant militaires qu'humanitaires, sur les modalités d'accueil des

Plus que jamais, nous voulons souligner que le multilatéralisme est un outil de conquête de la paix et du progrès de l'ensemble des peuples du monde. Mes chers collègues, je veux dire au nom de mon groupe, au nom du parti qui est le mien, comme sénateur socialiste comme citoyen, qu'avant toute considération, à l'instar de tous les Français, nous sommes républicains : nous croyons à la force, à la sagesse, à la beauté de la République, ce projet de fraternité universelle que la Nation s'est choisi il y a plus de deux siècles et auquel elle a régulièrement démontré son attachement, notamment lors de la Seconde Guerre mondiale. Plus que jamais, dans la tempête et devant les incertitudes, nous affirmons que nous défendrons cette flamme, car elle est un phare dans le monde. En ce sens, sans rien concéder ni de la richesse de nos différences ni de la puissance du débat démocratique, nous prenons l'engagement de travailler avec détermination et vigilance dans l'unité républicaine pour parvenir à passer tous ensemble cette terrible épreuve pour la France, pour l'Europe et pour le monde. Mes chers collègues, l'Ukraine nous oblige, l'Ukraine martyre mène un combat à mort pour la liberté, non seulement la sienne mais aussi la nôtre. Permettez-moi de saluer ici l'extraordinaire bravoure et, peut-être, le sacrifice suprême du président Zelensky, qui, cette après-midi, dans un échange avec les parlementaires européens, a proclamé : « Ne nous lâchez pas, la lumière doit vaincre l'obscurité ! » Gloire à l'Ukraine

Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, madame la ministre, messieurs les ministres, mes chers collègues, au sixième jour de ce terrible conflit, alors que les chars russes sont aux portes de Kiev, mes premières pensées vont au peuple ukrainien et à ses dirigeants, qui font preuve d'un courage et d'un héroïsme forçant l'admiration. Mes pensées vont également à nos compatriotes, pris au piège de la guerre aux portes de l'Europe. Après avoir annoncé, le 21 février, la reconnaissance de l'indépendance des territoires séparatistes du Donbass, Vladimir Poutine a commis l'irréparable en pénétrant en Ukraine à l'aube du 24 février, réduisant à néant les accords de Minsk, qui portaient l'espoir d'une solution diplomatique. Pis, il se justifiait en réaffirmant sa volonté de « démilitariser » et de « dénazifier » le pays, tout en le protégeant d'un « génocide » programmé Cette guerre est décidément celle de la désinformation et de l'image, une guerre de l'intox visant à déstabiliser une armée sur le plan psychologique. Mais tout cela était sans compter sur la capacité de résistance de l'armée ukrainienne, sans compter sur la détermination du président Volodymyr Zelensky, sans compter sur la capacité de réaction unifiée de l'Europe. Le délire paranoïaque de Vladimir Poutine l'a amené à justifier cette intervention militaire en invoquant l'article 51 de la Charte des Nations unies relative à la légitime défense. « La sécurité absolue d'un acteur implique l'insécurité absolue de tous les autres », écrivait Henry Kissinger en parlant de l'URSS. Cette phrase est plus que jamais d'actualité et résume à elle seule la schizophrénie de Vladimir Poutine. Après l'Ukraine, quel sera le prochain pays à faire l'objet des velléités du dirigeant russe ? La Moldavie ? La Géorgie ? Le maître du Kremlin, depuis son accession au pouvoir, n'a cessé de déclarer que le droit de sécession des quinze républiques de l'ex-URSS était une erreur historique et que la dislocation du bloc socialiste était la plus grande catastrophe géopolitique du XX siècle. Comment un homme seul peut-il décider du destin de tout un peuple ? En bafouant les règles du droit international, Vladimir Poutine s'est isolé du reste du monde. Face à la résistance ukrainienne et à la détresse de toute une population, l'Occident a retrouvé l'unité qui lui a longtemps fait défaut. En quelques heures, l'Europe de la défense a pris forme afin de répondre à la plus abjecte des provocations, certains pays allant même jusqu'à sortir de leur neutralité en appliquant les propositions de sanctions ou en proposant la fourniture d'armes létales. Alors oui, les sanctions économiques étaient nécessaires et amplement justifiées, et constituent un premier niveau de réponses. Le deuxième volet de mesures de rétorsion décidées ce week-end paraît totalement adapté à la situation et à son aggravation la fermeture de l'espace aérien de l'Union européenne à la Russie, l'interdiction de la diffusion des médias d'État russes ou encore l'isolement du réseau bancaire Swift des marchés internationaux. Pour autant, cela suffira-t-il à dissuader Vladimir Poutine de mener une offensive destructrice sur l'ensemble du territoire ukrainien ? Nous n'en avons aucune certitude et il est permis d'en douter. À l'issue des sommets européens, des réunions du G7 et de l'OTAN, le chemin du dialogue reste possible. Même si, au sixième jour de cette offensive, l'intensité des combats ne faiblit pas, nous devons conserver et privilégier la voie diplomatique pour résoudre le conflit. Les évènements de ces derniers jours marquent un tournant historique et plongent l'ensemble du continent européen dans l'incertitude. Pour autant, monsieur le Premier ministre, ne laissons pas croire à l'Ukraine qu'elle pourrait demain adhérer à l'Union européenne par le biais d'une procédure simplifiée qui n'existe pas. Au-delà du drame humain qui se joue en ce moment, et sur lequel reviendra ma collègue Nadia Sollogoub, présidente du groupe d'amitié France-Ukraine, nous devons également nous préparer au risque et aux dommages collatéraux engendrés par cette crise majeure. Un manque d'approvisionnement et une flambée des prix sont à craindre sur bon nombre de marchés internationaux de matières premières, tels que ceux du blé, du maïs, du gaz ou du pétrole. La volatilité des prix sur le marché de l'énergie sera particulièrement inquiétante. La question des stocks actuels et les perspectives quant à nos approvisionnements en minerais et en métaux risquent d'être encore plus compliquées. Je pense notamment au palladium, au titane, indispensables à nos industries aéronautiques et de l'armement, ou encore au nickel, nécessaire à la fabrication de nos batteries. Ces heures sombres démontrent que les vingt-sept pays de l'Union européenne sont en mesure de formuler des réponses communes, fortes et rapides, qui doivent nous amener également à renforcer plus encore nos partenariats européens et transatlantiques afin d'assurer la sécurité de nos territoires et de nos alliés. alliés. Personnellement, je suis persuadé que la solution viendra du peuple russe, en contradiction avec la vision paranoïaque et velléitaire du dictateur du Kremlin. Alors oui, monsieur le Premier ministre, l'heure est à l'unité et à la solidarité. Vive l'Ukraine et vive la France

Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, madame la ministre, messieurs les ministres, mes chers collègues, si le peuple ukrainien et son président suscitent autant d'émotion, autant d'admiration, c'est parce qu'aujourd'hui, par leur courage, par leur détermination sans limite, ils ne défendent pas seulement leur nation et leur territoire : ils incarnent la volonté farouche de résister à l'arbitraire, à la soumission, à l'agression. Ils aspirent à la souveraineté, à la liberté, à la démocratie ; ils défendent ces valeurs qui sont aussi les nôtres au prix du sacrifice ultime. La résistance de ce peuple et de ces soldats aguerris face aux offensives militaires russes nous inspire. À ce titre, nous leur devons un soutien sans faille, ferme et déterminé, par des actes qui leur permettront de résister et de garder espoir, comme vous l'avez très bien dit, monsieur le Premier ministre. Je veux dire ici au président Zelensky tout notre respect, toute notre admiration. Il incarne le chef de guerre que tant de peuples rêvent d'avoir : héroïque, inflexible au milieu de ses hommes et prêt à périr pour son peuple et pour notre paix à tous. Ce jeudi 24 février 2022, l'Europe s'est brutalement réveillée dans une ère de guerre. On le redoutait. Le Président de la République et le Chancelier allemand ont tout tenté, par la négociation, par la médiation, pour l'éviter. Ce scénario du pire s'est finalement réalisé parce que le président russe, porté par son ivresse de puissance, a décidé de faire fi du droit international, des principes de souveraineté et d'intangibilité des frontières, pour agresser militairement un État souverain, pour envahir l'Ukraine, alors même que la Russie n'était ni agressée ni menacée. Cette tragique bascule nous ramène à nos souvenirs les plus effroyables de la guerre froide. Aux quatre coins de l'Ukraine, ce sont désormais les sirènes d'alarme antiaérienne, les tirs, les explosions des bombes, les victimes civiles et militaires qui jalonnent les jours et les nuits. Voilà deux heures à peine, une frappe russe a touché la tour de la télévision à Kiev. À elle seule, cette frappe a visé ce qui est de plus cher à nos yeux : la liberté d'expression et la liberté d'information. À cette heure, j'ai aussi une pensée pour nos ressortissants sur place. Je remercie l'équipe de notre ambassadeur, Étienne de Poncins, qui poursuit l'accompagnement de nos concitoyens. Mes chers collègues, avec le recul, que l'allocution télévisée du président russe annonçant sa reconnaissance des républiques autoproclamées du Donbass, quatre jours avant le début de cette guerre, constituait les prémices de sa réelle intention. longues minutes durant lesquelles nous avons assisté à une réécriture surréaliste de l'Histoire, un discours composé de fausses accusations contre l'Ukraine. Les mots étaient minutieusement choisis pour poser les premières pierres de son mensonge. En l'espace de quelques jours à peine, les masques sont tombés, d'hallucinants motifs sont venus justifier son passage à l'acte. Qui peut croire qu'un « génocide » est en cours en Ukraine et qu'une « dénazification » est nécessaire pour la survie de la Russie ? Dimanche, la pression a atteint son paroxysme lorsque, face à des résultats militaires limités et à la multiplication des gestes de soutien envers Kiev, Vladimir Poutine, dans une démonstration désinhibée de puissance, a déclaré mettre les forces de dissuasion de l'armée russe en régime spécial d'alerte au combat. Comment la Biélorussie peut-elle continuer à être complice d'une telle escalade mortifère ? Vladimir Poutine voulait recréer l'URSS ; il a fait l'unanimité contre lui, il a réveillé l'Europe, il a redonné tout son sens à l'OTAN. Ensemble, nous avons déconnecté notre ciel européen. Nous faisons le choix d'accélérer la lutte contre la désinformation russe, au point d'aboutir à l'interdiction totale de deux outils de propagande du Kremlin, RT et Sputnik, sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne. J'appelle les réseaux sociaux à se battre à nos côtés. À l'unisson des autres pays occidentaux, nous avons déployé d'innombrables sanctions économiques, d'une force de frappe sans précédent : sanctions contre les réserves en devises de la banque centrale de Russie ; exclusion de plusieurs banques russes du réseau interbancaire Swift. Et bien d'autres encore. La démarche est sans équivoque provoquer une véritable onde de choc dans la société russe pour pousser les citoyens à remettre en question la propagande du Kremlin. Les premiers résultats sont là. Ensemble, faisons le choix de l'unité et de la solidarité face à l'impact humanitaire et à la crise migratoire que cette guerre entraîne aujourd'hui. Pour la première fois, nous avons enclenché le dispositif de protection temporaire automatique, avec des mesures pour répartir l'accueil des réfugiés entre les pays membres. Je saisis cette occasion pour remercier nos communes, nos intercommunalités, nos villes, nos régions, mobilisées pour accueillir des réfugiés ou pour contribuer à l'aide d'urgence en faveur du peuple ukrainien. Je remercie les associations et je remercie nos concitoyens leur élan de générosité fait l'honneur de la France. Enfin, la nécessaire autonomie stratégique de l'Union européenne, évoquée par le Président de la République dès le discours de la Sorbonne en 2017- vous l'avez rappelé, monsieur le Premier ministre -, n'a jamais connu un écho aussi retentissant. Pour la première fois de son histoire, l'Union européenne a annoncé débloquer 450 millions d'euros pour acheter des armes létales destinées à être livrées aux forces armées ukrainiennes, ainsi que du carburant. La Suède et l'Allemagne rompent avec leur doctrine selon laquelle elles ne livrent pas d'armes létales à un État en guerre. L'Allemagne va plus loin encore : ce dimanche, devant le Bundestag, le chancelier Scholz a opéré un virage à 180 degrés dans la posture militaire du pays en annonçant une hausse des dépenses de défense, qui dépasseront 2 % de son PIB annuel, et la création d'un fonds spécial de 100 milliards d'euros pour renforcer ses capacités de défense. C'est un tournant historique, c'est un tournant majeur. Même la Suisse sort de sa neutralité ! Nos actions, nos sanctions et notre détermination sont dictées par une unique raison : la paix. Je veux saluer ici la démarche du Président de la République, qui a toujours cru à la diplomatie et qui poursuit un dialogue avec lucidité, fermeté et courage. Monsieur le Premier ministre, nous sommes conscients de l'impact que nos sanctions pourraient aussi avoir sur notre quotidien. Nous y sommes prêts au nom de notre sécurité collective et de la paix, parce que nous savons pouvoir compter sur le soutien du Gouvernement pour établir un plan de résilience qui soit à la hauteur. Et vous pourrez compter sur nous pour identifier les mesures qui aideront au mieux nos concitoyens. Nous affronterons ensemble les difficultés : il y va de la force de nos démocraties et de l'unité de l'Europe. Reculer devant le coût des sanctions, c'est s'exposer à devoir payer un prix infiniment plus lourd si le président russe atteint son objectif. Car d'autres bruits de bottes, en d'autres points du monde, n'attendront plus que le moment opportun pour se faire entendre.

communiste républicain citoyen et écologiste. Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, madame la ministre, messieurs les ministres, mes chers collègues, la guerre déclenchée par Vladimir Poutine contre l'Ukraine le 24 février est inacceptable, elle est irresponsable, elle plonge le peuple ukrainien dans un cauchemar insoutenable, elle menace la sécurité de l'Europe et du monde. Le risque d'une escalade incontrôlable augmente chaque jour. La situation est donc d'une extrême gravité. Quelle que soit l'opinion que l'on ait sur les causes de cette entrée en guerre de la Russie- j'y reviendrai -, je veux redire ici la condamnation totale qui est la nôtre : cette guerre est un crime contre la souveraineté d'un État, l'Ukraine, un crime contre le droit international, un crime contre la paix. Rien ne peut excuser le sort infligé à des millions d'Ukrainiens aujourd'hui sous les bombes ou sur les routes de l'exode, dont nous sommes solidaires. Dans un monde si interdépendant, cette guerre est un échec pour tous et un échec pour la sécurité collective de l'Europe. Elle montre les limites dangereuses atteintes par la militarisation des relations internationales et son cortège de discours guerriers, de haine et de nationalisme. Pour toutes ces raisons, parce que cette guerre est illégitime et illégale, parce qu'elle est inhumaine pour le peuple ukrainien, parce qu'elle menace la sécurité du monde, parce qu'elle risque de nous entraîner vers l'irréparable, la première des exigences que nous clamons haut et fort est celle d'un cessez-le-feu immédiat,

Le vote de l'assemblée générale extraordinaire en cours à l'ONU sera un moment important. Faisons entendre les mobilisations citoyennes qui exigent partout le cessez-le-feu et la paix. Saluons les manifestations courageuses en Russie en demandant la liberté des opposants à cette sale guerre. Nous ferons tout, en ce qui nous concerne, pour encourager les mobilisations populaires pour la paix. Les sanctions internationales contre le régime de Poutine peuvent participer à cette pression, à condition qu'elles frappent juste. Il s'agit pour nous non pas de mettre à genoux un peuple, mais d'isoler un pouvoir oligarchique, autoritaire, fauteur de guerre. Le risque est grand, de punir les peuples, en Russie et ailleurs, alors que les sanctions doivent viser le cercle du pouvoir impliqué dans les décisions guerrières et les oligarques qui pillent leur pays sans vergogne, avec la complicité tacite- et depuis bien longtemps -du monde de la finance internationale. Les tergiversations sur Swift montrent d'ailleurs le degré d'intimité qui règne dans la haute finance et les paradis fiscaux. Retenons au passage qu'il est donc possible, quand on en a la volonté politique, de cibler les flux financiers au plus haut niveau. Autre urgence : tout doit être fait pour renforcer l'aide humanitaire et sécuriser son accès aux zones de conflit, conformément au droit humanitaire international, avec la livraison de matériel de protection, l'accueil des réfugiés

même si le tri ethnique que semblent vouloir organiser la Pologne et la Hongrie avec la complicité de l'Union européenne est parfaitement indécent. L'Union africaine s'en est émue hier : on ne trie pas les victimes des guerres Les livraisons d'armes sont l'autre sujet brûlant. Face à l'agression russe caractérisée, qui oserait dénier à l'Ukraine le droit de se défendre ? La France parle d'aider à renforcer ses moyens de défense, mais on entend aussi parler d'avions de chasse, ce qui pourrait impliquer directement ou indirectement le système de l'OTAN. Le Parlement doit être clairement informé et connaître avec précision ce qui a été livré et ce qui sera livré. Son contrôle sur ces évolutions rapides est essentiel. J'entends des hourras saluer le soudain emballement militaire de l'Union européenne et l'annonce d'un réarmement de l'Allemagne à hauteur de 100 milliards d'euros, le double de notre budget militaire. La gravité des enjeux devrait nous inciter à plus de clairvoyance et de lucidité. Il s'agit là de questions hautement inflammables. La frontière est fragile vers une escalade entraînant dans la guerre des pays européens membres de l'OTAN, une escalade aux conséquences alors incalculables. La mise en alerte de la force de dissuasion russe par Vladimir Poutine est, dans ce contexte, parfaitement irresponsable. Toutes les puissances nucléaires, parmi lesquelles figure la France, ont l'immense responsabilité de ne pas entraîner le monde dans cette folie. À ce sujet, la déclaration de Bruno Le Maire, qui parle de « guerre totale à la Russie », jette dangereusement de l'huile sur un feu déjà brûlant. Tout n'a pas été fait pour éviter la guerre. Des efforts pour une désescalade ont été engagés, mais tout n'a pas été fait dans ce sens, ou bien trop tardivement. Aujourd'hui, la guerre ne doit pas éteindre les efforts de paix ; elle doit au contraire les renforcer. les renforcer. J'entends la voix des boutefeux nous dire qu'il faut oublier tout cela, que seul importe d'armer l'Ukraine. Mais la guerre, c'est le peuple ukrainien qui en est la première victime Le cessez-le-feu, l'arrêt des bombardements, la reprise de discussions de paix respectant la souveraineté de l'Ukraine doivent rester la colonne vertébrale de l'action de la France. La paix est plus que jamais une affaire de sécurité globale et collective. La guerre en Ukraine nous dit combien la militarisation des relations internationales a atteint sa cote d'alerte. Dès la décennie 1990, après la dissolution du Pacte de Varsovie, des opportunités historiques se présentaient pour construire un monde débarrassé de l'affrontement des blocs, ouvrant la voie à un désarmement massif. C'est le contraire qui a été fait Tandis que les oligarques pillaient la Russie sous le regard complice de multinationales à l'affût de leur part du gâteau, la seule logique à l'oeuvre fut celle de l'extension de l'OTAN et de l'hégémonie mondiale. Après l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir, les États-Unis ont poussé les feux de cette confrontation et les Européens n'ont jamais trouvé les voies d'une parole unie et indépendante pour ouvrir le chemin du dialogue avec la Russie sur ce qu'Emmanuel Macron appelait en 2018 « une nouvelle architecture de sécurité européenne », ou sur ce que nous appelons, pour notre part, « une initiative multilatérale pour un nouveau traité paneuropéen de paix et de sécurité La Russie s'est enfoncée dans cette logique guerrière de confrontation, singulièrement depuis 2014 et l'annexion de la Crimée jusqu'à cette guerre dramatique en Ukraine. il faut le dire, jamais l'occasion ne fut saisie pour ouvrir sérieusement de réelles voies de négociations, laissant la confrontation et la force seules s'exprimer. Vingt ans d'obsession otanienne pour le surarmement, vingt ans de réarmement russe, vingt ans d'exacerbation des nationalismes : le bilan est désastreux. Que de temps perdu, qu'il faudra maintenant regagner en faveur de la paix ! Alors oui, même au coeur de ce terrible orage de bombardements, la paix doit rester notre projet politique. La paix, et non pas l'équilibre de la terreur ou la confrontation des puissances. La paix pour l'Ukraine, avec le cessez-le-feu immédiat et le départ des troupes russes. La paix pour la Russie, qui doit trouver avec l'Europe les conditions d'une sécurité sans l'OTAN à ses portes. Même quand il paraît si étroit, un chemin existe toujours pour le dialogue.

La paix pour tous les Européens, qui doivent assurer leur sécurité souverainement, dans le respect mutuel des États, sans la tutelle américaine otanienne. La paix par le désarmement nucléaire et conventionnel multilatéral. La paix partout dans le monde, en Afrique, au Moyen-Orient, avec la fin des opérations militaires extérieures. Oui, mes chers collègues, comme l'a déclaré le secrétaire général des Nations unies, le 18 décembre dernier, en recevant la Lampe de la paix de saint François

Monsieur le président, Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, madame la ministre, messieurs les ministres, mes chers collègues, en 1991, la chute de l'URSS et du rideau de fer annonçait pour beaucoup la fin de l'Histoire et le triomphe à venir d'un modèle universel de démocratie libérale. Malheureusement, trente ans plus tard, comme si la guerre de Yougoslavie n'avait pas suffi, le nationalisme fait son retour tragique aux portes de l'Union européenne en charriant son lot de désespoir et de désolations. L'invasion injustifiée et inqualifiable de l'Ukraine par l'armée russe sonne bien comme un tragique retour en arrière. De 2014 à 2022, d'une conférence de Munich à l'autre, la séquence diplomatique, beaucoup plus longue en réalité que ce qu'en a perçu l'opinion publique, a laissé la place aux armes. La guerre est au coeur de l'Europe et menace l'ordre international établi depuis la Seconde Guerre mondiale, fondé sur le respect du droit international et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Au nom du RDSE, je tenais à exprimer notre solidarité sans réserve à l'égard du peuple ukrainien, qui se bat pour sauver la souveraineté de son pays et sa liberté. Je salue son courage, ainsi que celui du président Zelensky, demeuré au coeur de la capitale assiégée et présent aux côtés de ses soldats et de la population. J'ai également une pensée pour les Ukrainiens de France, qui s'inquiètent pour leurs proches. Enfin, mon groupe souhaite que l'Union européenne accueille dans les meilleures conditions les réfugiés qui affluent. Il va de soi que c'est un devoir moral, mais aussi une nécessité politique pour montrer que notre vision de ce qu'est une société est à l'opposé du projet mortifère qui se déploie en Ukraine. Je pense également au peuple russe, qui va payer le prix de l'isolement politique et économique. Il faut rappeler que beaucoup de Russes, soit par peur, soit par résignation, soit par un patriotisme mal alimenté, ne font que subir la posture martiale de leurs dirigeants, bien aidés- il faut le souligner -par une propagande intérieure très efficace. La situation des États baltes, de la Pologne et de la Roumanie, qui sont nos alliés et amis au sein de l'OTAN, doit aussi retenir toute notre attention. Nous savons que le chef de l'État leur a donné tous les gages de notre soutien. Je pense aussi à la situation de la Moldavie, dont une partie du territoire est occupée par l'armée russe, et qui ne doit pas devenir la prochaine visée de l'expansionnisme de Moscou. Je pense également à nos amis suédois et finlandais, nommément menacés par le chef de l'État russe. Enfin, je n'oublie pas nos concitoyens français, qui, après deux ans de guerre contre un virus, aspiraient au retour à une vie normale. Ils observent avec incrédulité et angoisse la guerre à quelques heures d'ici, sans savoir quand et comment elle s'arrêtera. En attendant, nous devons tenir un langage de vérité. Le Président de la République s'est exprimé en ce sens. Il faut nous préparer à parer à toutes les situations, y compris les pires.

Les démocraties ne sont évidemment pas prêtes à s'engager dans un conflit frontal. La dissuasion nucléaire joue pleinement son rôle, mais montre aussi ses limites. Dans ces conditions, sanctionner l'économie russe et s'attaquer aux oligarques semblent constituer pour le moment le meilleur outil de pression contre le régime russe et son vassal biélorusse, même si, encore une fois, la population sera la première à en souffrir. Cependant, à court terme, cette stratégie sera coûteuse pour les Ukrainiens, qui vont devoir résister en espérant tenir. Le soutien matériel et humanitaire doit être amplifié autant que possible. La France s'en honore, comme tous ses partenaires. partenaires. La décision historique de l'Union européenne d'envoyer du matériel militaire létal permettra peut-être, à plus long terme, de catalyser la formation d'une Europe enfin souveraine sur le plan stratégique et militaire. La décision de l'Allemagne de se réarmer montre aussi que, paradoxalement, la décision d'envahir l'Ukraine coûtera à la Russie, sur le long terme, la formation d'un bloc ouest européen plus uni et plus puissant.

Cependant, le renoncement est très vite apparu inenvisageable. Le groupe du RDSE soutient donc sans réserve la politique de sanctions décidée conjointement par les États-Unis, l'Union européenne et de nombreux autres pays du monde. Les premiers effets peuvent déjà être mesurés. il est évidemment trop tôt pour en tirer des conclusions, car le géant russe peut aussi se tourner vers son partenaire chinois- bien qu'il n'existe pas d'amis en géopolitique, mais seulement des intérêts convergents. convergents. L'activité diplomatique doit, bien entendu, se poursuivre. Le maintien d'un dialogue, certes exigeant, reste la clef de la résolution du conflit. Ce dialogue, même biaisé, existe bien : entre les belligérants, mais aussi entre l'Union européenne et le dirigeant russe, hier encore par la voix du Président de la République. Toutes les initiatives en ce sens doivent être encouragées et soutenues. Néanmoins, à ce jour, les conditions d'un règlement du conflit posées par le président russe demeurent inacceptables. Au sein de la communauté internationale, il faut continuer à isoler Moscou. La Chine et la Turquie ont émis des signes de retenue qui doivent être préservés. Je rappellerai ainsi un principe formulé par le général et théoricien militaire prussien Clausewitz : « La guerre n'est pas seulement un acte politique, mais un véritable instrument de la politique, une poursuite de relations politiques, une réalisation de celles-ci par d'autres moyens. » Vladimir Poutine sait parfaitement entremêler diplomatie et actes de guerre. Après tout, le conflit d'aujourd'hui n'est que la continuation de ce qui se passe au Donbass et en Crimée depuis au moins 2014. Bien sûr, il est toujours facile de réécrire l'Histoire. Oui, peut-être, une fois le mur tombé, aurait-il fallu créer une véritable organisation de la sécurité en Europe qui n'aurait pas constitué un épouvantail pour le Kremlin. Mais n'inversons pas les responsabilités Oui, notre main a sans doute tremblé un peu lorsque les troupes russes sont entrées en Transnistrie en 1992, en Géorgie en 2008 ou ont annexé la Crimée en 2014. Oui, il est possible que nous ayons sous-estimé le rêve poutinien d'une grande Russie, alors même que plusieurs indices étaient présents, encore récemment au travers de l'allégeance du président biélorusse Loukachenko. Quelle que soit l'histoire, le temps n'est plus au regret, d'autant qu'il est difficile de savoir ce qui aurait pu arrêter le dirigeant russe dans sa volonté d'expansion et d'hégémonie. Le discours du 21 février dernier n'était ainsi qu'une réécriture fallacieuse de l'histoire de l'Ukraine, servant à justifier l'invasion. Mes chers collègues, pour conclure, dans ce climat empreint d'une extrême gravité, je souhaiterais malgré tout souligner un point positif. Il s'agit de la remarquable unité que l'Union européenne a manifestée dans cette épreuve Après la solidarité sanitaire et la solidarité budgétaire, la solidarité est au rendez-vous pour assurer notre sécurité collective. Espérons que, conjuguée à l'appui de nos nombreux alliés, cette unité pourra contribuer à sauver la paix, la liberté et l'indépendance de l'Ukraine.

Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, l'invasion de l'Ukraine pourrait bien être le premier clou sur le cercueil de la dictature de Poutine, comme l'invasion de l'Afghanistan fut le premier clou sur le cercueil de l'Union soviétique. Poutine est fou comme le sang est rouge. Ce n'est pas une insulte, c'est un diagnostic. Le discours sépulcral du 21 septembre ne laisse aucun doute : c'est un paranoïaque doublé d'un mythomane. Plus il élimine toute contradiction, plus il échappe à la réalité, au profit de son idée fixe et funeste : se venger de la chute de l'URSS. Comme beaucoup de dictateurs, ce Caligula botté souffre d'une autre infirmité.

Néron se faisait raser par ses filles de peur d'être égorgé, Staline faisait goûter ses aliments, lui, chef de la deuxième force nucléaire au monde, qui se fait filmer dans de fausses chasses à l'ours, pétoche devant le virus comme un matamore fuyant devant une souris. En face de lui, un homme, debout : Zelensky. Lorsqu'on ignore la réalité, elle se venge. Poutine voulait diviser l'Europe, il la cimente. Il voulait ridiculiser l'OTAN, il la retrempe. humilier les États-Unis, il ressuscite Biden après Kaboul. Il voulait rallier à lui les régimes autoritaires ; la Chine s'inquiète, la Turquie montre les dents, et le Kazakhstan refuse l'envoi de ses soldats. Il pensait prendre l'Ukraine en trois jours, il est embourbé pour longtemps. Confiné dans son bunker, il n'a pas vu le monde changer. Il se croit encore au temps où ses complices du KGB et du mataient par des chars la Hongrie ou la Tchécoslovaquie, et où lui-même rasait Grozny à l'abri des caméras. Il n'a pas compris que les images des smartphones faisaient le tour du monde en une seconde et qu'en 2022 personne, pas même les Russes, n'était prêt à accepter les bombardements de Kiev et les morts. S'il en est arrivé là, c'est en partie à cause de nos propres lâchetés. L'invasion de la Géorgie, l'annexion de la Crimée, le Donbass, la Transnistrie, les crimes contre l'humanité commis en Tchétchénie ou en Syrie, les centaines d'assassinats et les milliers d'emprisonnements en Russie même : tout cela, nous l'avons laissé faire. ont été prononcés à l'ONU sur les droits de l'homme et le droit international, et puis, circulez, il n'y a rien à voir ! Ce n'est pas seulement par lâcheté que nous n'avons rien fait. C'est parce que les démocraties ont en leur sein une cinquième colonne, le plus souvent soudoyée par le Kremlin, qui reprend mot à mot sur les réseaux antisociaux, au moyen de milliers de faux comptes, de trolls et de pilotés depuis Moscou, sur les radios et télévisions de RT, Sputnik et, hélas !, d'autres encore, la propagande de Poutine : l'Ukraine n'existe pas, elle est dans la sphère russe, ses dirigeants sont des nazis. Vladimir Zemmour, Joseph Vissarionovitch Mélenchon et Anastasia Le Pen sont depuis longtemps les généraux en chef de cette cinquième colonne. Mais leurs dernières déclarations atteignent des sommets. Mélenchon a ainsi déclaré le 18 janvier dernier : « Qui ne ferait pas la même chose avec un voisin pareil, un pays lié à une puissance qui les menace continuellement ? : « Mon point de vue sur l'Ukraine coïncide avec celui de la Russie. » Quant à Zemmour, il a affirmé : « Il faut arrêter de faire de Poutine l'agresseur, c'est Poutine l'agressé. Poutine est l'allié qui serait le plus fiable.

Le pire, c'est Zemmour, le trois fois condamné pour racisme, qui crache sur les résistants ukrainiens et sur les réfugiés, et qui donne des leçons de patriotisme, lui qui, après s'être soustrait au service militaire, n'a pas hésité à se rendre samedi sur le plateau des Glières. Ses propos souillent les tombes des maquisards. Ces paillassons de Poutine, après en avoir été les caniches, sont candidats à la Présidence de la République. Ils ont condamné le dictateur du bout des lèvres, mais leurs trolls inondent les réseaux de messages à sa gloire et leurs députés européens ont refusé de voter l'aide à l'Ukraine. Pendant des années, nous avons tenté de faire comprendre qui était Poutine. Nous étions trop peu nombreux face aux idiots utiles de l'Europe. L'Allemagne s'est mise dans les griffes de l'ours et de son gaz l'incroyable erreur de céder aux Verts sur le nucléaire. En France, le fond de l'air, fait d'un gaullisme du pauvre qui n'a rien à voir avec le gaullisme et d'un antiaméricanisme héritier de la vieille droite anti-anglo-saxonne et de la vieille gauche anticapitaliste, conduit certains à prêcher l'équidistance entre l'Amérique et la Russie- et, demain, entre l'Amérique et la Chine -, sans comprendre qu'il y a d'un côté le camp de la démocratie et de l'autre celui des dictatures. Trop peu nombreux, nous étions par là même trop faibles. Le 24 février 2022 restera dans l'Histoire comme le jour prodigieux du grand basculement. Le plus grand succès de Poutine, c'est de nous avoir ouvert les yeux. Nous nous sommes réveillés bien tard, mais nous nous sommes réveillés Pour la première fois, nos sanctions sont plus que des coups de griffe. Elles comprennent le blocage des réserves de la banque centrale, la déconnexion du système Swift, l'arrêt de Nord Stream 2, la saisie des avoirs des corrompus, la fermeture des espaces aériens, le bonheur de la livraison d'armes aux Ukrainiens par l'Allemagne elle-même- mouton devenu, non pas tigre, mais au moins lionceau- et, enfin, la chasse aux agents de désinformation. Voilà cinq ans que je demande la fermeture de RT, de Sputnik et de leurs satellites, cinq ans que l'on me répond que ce serait bafouer la liberté d'expression. On vient enfin de comprendre que les organes de propagande du FSB n'ont rien à voir avec la liberté d'expression. Mesdames, messieurs les dirigeants européens, permettez-moi d'ajouter à mes félicitations pour ces sanctions une supplique qu'elles soient précises, sans exception, efficaces, non contournables et prolongées, et surtout qu'elles soient rapides et accrues car les résistants ukrainiens, aussi héroïques soient-ils, ne tiendront pas longtemps par leurs seuls moyens. enfin qu'elles soient accompagnées du message clair selon lequel l'assassinat de Zelensky entraînerait une riposte bien plus massive encore. Quant à la cinquième colonne, elle va se déchaîner dans toute l'Europe pour relayer les menaces du tyran et expliquer que, comme vous êtes responsables de la guerre en Ukraine, vous serez responsables, demain, de la troisième guerre mondiale dont Poutine brandit la menace. Pour l'heure, autre miracle : personne n'y croit. Comment penser qu'un hypocondriaque qui s'ausculte toute la journée soit prêt à mourir sous les frappes ou à finir ses jours dans un abri antiatomique, comme Caïn dans son souterrain ? Lorsque nous aurons pris ces sanctions et que nous nous serons préparés à un long conflit- car cette guerre sera longue -, il nous faudra relever un autre défi, plus redoutable encore : celui du rétablissement de la puissance de l'Europe. L'Europe ne se fera qu'au bord du tombeau », disait Nietzsche. Ces propos étaient prophétiques, car l'Europe est née des charniers de la Seconde Guerre mondiale et n'a progressé qu'en surmontant ses crises. Celle du covid-19 a permis un pas de géant par la mutualisation des dettes du plan de relance. L'invasion sanglante de l'Ukraine a fait comprendre à tous, à commencer par les Allemands, ce que le Président de la République ne cesse d'expliquer depuis le début de son mandat : l'Europe ne sera jamais une puissance si ses États ne se réarment pas et si une défense commune ne voit pas le jour. Jamais Poutine n'aurait pu nous faire un meilleur cadeau. Pour l'heure, nous allons participer à cette guerre au moyen des mesures déjà prises, de notre unité avec nos alliés européens et américains, et de notre fermeté face au tyran qui s'est lancé dans une aventure sans issue. Toutefois, ce n'est pas nous qui allons la gagner. Les seuls qui peuvent la gagner, ce sont deux peuples. du peuple russe qui, pour la première fois, malgré une répression impitoyable et une propagande effrénée, est en train de comprendre que Poutine le conduit vers le gouffre. Le sursaut viendra-t-il de la rue, ou de quelques Brutus qui comprendront l'urgence d'agir avant qu'il ne soit trop tard ? Je ne sais. Cependant, le dénouement pourrait bien surprendre. surprendre. Ceux qui vont gagner cette guerre, ceux qui sont déjà en train de la gagner quel qu'en soit le coût, ceux qui nous donnent une grandiose leçon de courage, guidés par un président devenu en quelques jours un héros de la trempe d'un De Gaulle ou d'un Churchill, Volodymyr Zelensky, ceux qui vont gagner cette guerre, donc, ce sont surtout les membres du peuple ukrainien soudés contre Poutine et prêts au sacrifice pour défendre sa liberté- et la nôtre -, sa démocratie et les valeurs européennes qu'il partage. Puissions-nous les admirer, les acclamer, les soutenir et nous montrer dignes d'eux

Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, madame la ministre, messieurs les ministres, depuis six jours, nous vivons dans un état de sidération. La guerre est de retour en Europe, à l'initiative d'une grande puissance nucléaire qui déploie toutes ses capacités militaires contre un pays souverain. Nos pensées vont naturellement vers les Ukrainiennes et les Ukrainiens qui ont déjà perdu des proches, perdu des enfants, qui vivent en ce moment même la peur au ventre sous les bombes, sous les balles, au son des canons et des sirènes, ou qui ont tout abandonné derrière eux pour préserver leur vie et celle de leurs enfants. Ils et elles sont aujourd'hui les victimes d'une guerre d'agression indéfendable, d'une violation caractérisée du droit international d'un déploiement de violence commis par l'une des plus grandes armées au monde, sous la coupe d'un dictateur impérialiste et révisionniste qui refuse la simple existence de leur nation.

Volodymyr Zelensky, au courage et au sang-froid extraordinaires, et dont le monde entier connaît désormais le nom et le visage, vient nous rappeler une nouvelle fois que, bien plus que l'inverse, c'est l'Histoire qui fait les grands hommes. N'ayons pas peur des mots : le peuple ukrainien est aujourd'hui notre avant-garde sur le front oriental du combat pour la démocratie et la liberté. Cette sombre perspective a permis une prise de conscience généralisée de l'intérêt commun qui lie les démocraties et de la nécessité absolue, pour l'Europe, de devenir un acteur géopolitique. Nous saluons les décisions historiques des derniers jours. Le mot n'est pas galvaudé. Nous saluons l'action de la France et de l'Union européenne sous présidence française. Nous nous félicitons de l'extraordinaire unanimité des Vingt-sept. Sans le vouloir, Vladimir Poutine a ouvert la mer en deux et le chemin vers une Europe de la défense que les écologistes ont toujours défendue. Vladimir Poutine, qui depuis tant d'années joue de nos divisions, n'avait sans doute pas anticipé cet élan d'unité. Il s'était préparé à des sanctions économiques, mais vraisemblablement pas à des sanctions Ces sanctions n'épargneront pas le peuple russe, qui dans sa majorité n'a pas choisi cette guerre et qui est pétrifié par cette mise au ban des nations. Nous lui témoignons notre amitié et notre respect pour la mobilisation courageuse dont il fait preuve malgré les interdictions de manifester. Vladimir Poutine n'avait pas non plus anticipé la résistance militaire et l'héroïsme des Ukrainiennes et des Ukrainiens, qui ont empêché une prise rapide du pays. Si Kiev devait tomber entre les mains de Poutine, il ne pourrait maintenir son contrôle sur une population éprise de liberté. On n'occupe pas un pays contre son peuple. Nous n'en sommes cependant pas là encore. L'urgence est de venir en aide à la résistance ukrainienne. Nous approuvons le soutien financier, opérationnel, humanitaire et les livraisons d'armes que la France, l'Europe et nos partenaires transatlantiques lui apportent,

L'urgence est aussi de venir en aide aux réfugiés qui fuient l'Ukraine par millions. À ce titre, nous saluons la volonté de la présidence française de proposer jeudi prochain au Conseil de l'Union européenne l'activation de la directive relative à des normes La puissance publique doit faciliter le transit de celles et ceux qui veulent rejoindre l'ouest de l'Europe. Alors que l'Union africaine s'inquiète de la situation des ressortissants africains, dont certains seraient bloqués à la frontière par les autorités polonaises, et alors qu'un discours nauséabond s'installe doucement, visant à qualifier les réfugiés selon la couleur de leur peau ou leur religion, je veux rappeler ici avec force qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais réfugié. Toute personne, quelle que soit sa nationalité, a le droit de quitter un pays en guerre, et nous avons le devoir de l'accueillir. Aussi, nous demandons à la présidence française de faire preuve de la plus grande vigilance sur la situation aux frontières orientales de l'Union européenne et d'obtenir des garanties des pays concernés. Monsieur le Premier ministre, nous saluons- une fois n'est pas coutume -la démarche de transparence et de concertation que vous entreprenez malgré la complexité de la situation, et que nous espérons durable. Cette crise conforte notre rapport au monde et à l'Europe, et notre attachement à la liberté et à la démocratie. Le chemin de la paix est, hélas !, encore long, mais il passera inévitablement par une Europe unie, plus intégrée, capable de créer par la voie diplomatique les conditions d'un avenir pacifique et la sauvegarde de l'intégrité de la nation ukrainienne.

que ce n'est pas en jetant de l'huile sur le feu que l'on arrive à régler les problèmes. J'ai entendu un certain nombre de discours.

Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, madame la ministre, messieurs les ministres, mes chers collègues, les couleurs de l'Ukraine sont le bleu d'un ciel d'azur sur l'or des champs d'une terre fertile. Nous pourrons désormais y ajouter la trace indélébile du sang versé par un peuple héroïque qui tente, heure par heure, de résister à l'invasion de l'armée russe. Je vous parle ce soir avant tout en tant que citoyenne, une citoyenne française fière d'appartenir au continent européen. Je vous parle également en tant que présidente du groupe d'amitié France-Ukraine. En temps normal, l'amitié entre deux pays doit être le terreau de relations culturelles, économiques, commerciales et bilatérales qui croissent et prospèrent. En temps de guerre, l'amitié entre deux pays, ce sont les angoisses, les nuits blanches, les colonnes de réfugiés, les nouvelles auxquelles on ne peut pas croire, le décompte des victimes et la douleur de l'impuissance. Alors que d'immenses convois militaires convergent vers Kiev et que les missiles pleuvent sans cesse, l'urgence est d'obtenir une trêve, et une évacuation humanitaire. Les civils, femmes et enfants essentiellement, tentent de fuir, malgré la dangerosité du voyage. Les routes sont exposées aux frappes aériennes, constatées à neuf kilomètres de la frontière polonaise, nous a-t-on dit hier au Quai d'Orsay. Il y aurait eu ces jours derniers jusqu'à quatre-vingts heures d'attente pour entrer en Pologne, plus de trente heures pour la Moldavie. Alors que 650 000 civils ont déjà quitté l'Ukraine, ils pourraient être bientôt plus de six millions. Monsieur le Premier ministre, en plus de prendre en charge ces réfugiés qui arrivent de façon massive,

Les inquiétudes se portent aussi sur le ravitaillement. Bientôt, la capitale sera assiégée. Doit-on craindre un nouveau Sarajevo ? Hommes, femmes et enfants se retrouvent piégés, parmi lesquels un peu plus de 1 000 Français. Les cellules de crise réalisent un extraordinaire travail de contact individuel, de localisation, de recensement et de soutien, mais elles n'ont pas de solution à proposer, l'évacuation aérienne étant pour l'instant, hélas !, une hypothèse à écarter. Monsieur le Premier ministre, nous savons plus que jamais que les pires menaces prospèrent dans l'ombre. À cet égard, je souhaite exprimer une inquiétude particulière concernant la sécurité des installations nucléaires en Ukraine, M. l'ambassadeur d'Ukraine en France m'ayant alertée sur l'incapacité du pays à garantir le fonctionnement du site de Tchernobyl,

Danger à Kharkiv, danger à Kiev, danger sur les routes de l'exode, danger sur les sites sensibles : l'Ukraine n'est que danger et douleur. L'Ukraine n'est que courage. Face à l'ennemi, la pression massive d'une Europe unie et déterminée doit être absolue. Nous croyons en l'efficacité de cette stratégie, après avoir tant cru aux canaux diplomatiques qui, malgré tout, restent et doivent rester ouverts. Nous mesurerons dans les jours qui viennent l'impact de la rupture des échanges avec la Russie et, dans le même temps, les limites de nos fragilités et dépendances économiques et énergétiques. À court terme, il nous faudra nous adapter à des pénuries de matières premières, à un prix du carburant prohibitif, à des hausses de prix probablement difficilement supportables et à des pertes de marchés. La paix est à ce prix. Le groupe Union Centriste mesure tous ces enjeux et soutient fermement la politique nationale et européenne. Dans mes veines coule autant de sang russe que de sang ukrainien. Nous sommes nombreux dans ce cas. J'espère encore qu'un être humain ne puisse pas tuer son propre frère. Au péril de leur vie, près de 500 chercheurs et journalistes russes ont publié une tribune dans laquelle ils expriment leur protestation et exigent la paix. Cette guerre est injuste et absurde », disent-ils, « la guerre avec l'Ukraine est un pas vers le néant. » Il faut que Poutine, l'homme sans vérité, l'homme sans humanité, soit désormais un homme sans peuple et sans allié. qu'il soit seul, de plus en plus seul, et que ce soit son énorme et fatale fragilité. Le fil de l'histoire du peuple russe reprendra son cours. Faisons bien la différence entre le président Poutine et la nation russe qu'il tente de museler Nous sommes à l'heure des décisions collectives, qui doivent être à la mesure de l'immense leçon de courage que nous donne chaque Ukrainien, et en premier lieu le président Zelensky. « L'Ukraine se bat avec la certitude qu'elle défend le monde entier », nous a dit M. l'ambassadeur Vadym Omelchenko. Répondons-lui ici, dans ce même hémicycle, qu'il n'est pas seul, que l'Ukraine n'est pas seule, que le peuple ukrainien n'est pas seul., gloire à l'Ukraine ! La parole est

Territoires. Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, madame la ministre, messieurs les ministres, mes chers collègues, l'Ukraine n'a jamais menacé la Russie, encore moins les Russes. Ces Russes qui, par milliers, sont aujourd'hui détenus dans les geôles poutiniennes pour avoir courageusement marché dans les rues de Moscou et de Saint-Pétersbourg contre cette guerre infâme dans laquelle Vladimir Poutine les a entraînés.

C'est une guerre entre la volonté d'un peuple d'être libre et celle d'un tyran de l'en empêcher. Cette guerre n'est pas une guerre entre l'OTAN et la Russie. C'est une guerre entre la démocratie et la dictature, une guerre existentielle pour l'Europe entière, une guerre qui a réveillé la conscience de ce que nous sommes en tant que citoyens européens. Vladimir Poutine voulait affaiblir l'Europe : il a récolté sa force. Vladimir Poutine voulait diviser l'Europe : il a récolté sa plus puissante unité. Jamais on n'aura vu les Européens se mobiliser autant, dans toute l'Europe, pour crier leur refus de la brutalité, leur refus des chars et des missiles, leur solidarité sans équivoque avec le camp de la démocratie et de la paix. Jamais on n'aura vu les institutions européennes si unies et si efficaces, réagir si vite, si clairement et si massivement, ensemble. L'Europe renaît à Kiev. Elle renaît lorsque, au milieu des bombes, sous les tirs de missiles, Zelensky signe la demande d'adhésion à l'Union européenne. Ce faisant, il n'affirme pas seulement l'identité européenne de l'Ukraine : il affirme l'identité politique de l'Europe. Il rappelle pourquoi et contre quoi nous avons construit l'Europe. Il nous rappelle ce que nous sommes et ce que nous devons faire pour le protéger. Il nous rappelle que nous devons nous doter d'une politique de défense commune, arrimée à nos valeurs, et sortir sans attendre des énergies fossiles, ce qui implique

celles et ceux qui vivent dans les États dépendant encore massivement du gaz russe. C'est notre honneur de les assumer collectivement et de venir en aide, en Européens, à celles et ceux qui paieront le prix le plus fort pour protéger la paix de toutes et tous. Nous devons aux Ukrainiens, qui paient de leur vie la défense de nos valeurs, d'être à la hauteur du moment. Nous devons poursuivre avec eux la construction de notre projet commun : celui d'une Europe libre, d'une Europe de la solidarité et de la paix. La parole

Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, madame la ministre, messieurs les ministres, mes chers collègues, l'offensive russe contre l'Ukraine provoque une onde de choc, en Ukraine d'abord, où l'on déplore déjà tant de victimes civiles, mais aussi dans tout le continent européen. Renouant avec des heures sombres qu'on espérait révolues, l'Union européenne se trouve directement menacée à ses frontières par une Russie qui, après l'annexion de la Crimée en 2014, a décidé d'agresser l'Ukraine, ébranlant ainsi l'ordre international établi et menaçant la démocratie, la paix et la liberté, qui sont les valeurs fondatrices de l'Union européenne. Face à ce séisme, l'Union européenne a réagi rapidement et a fait preuve d'unité en adoptant des sanctions particulièrement sévères contre la Russie : gel des avoirs et interdiction de séjour pour les plus hauts dirigeants russes, y compris le président Poutine, suspension des vols vers la Russie, bannissement des médias d'État russes qui mènent des actions de désinformation en Europe et exclusion de plusieurs banques russes du système interbancaire international Swift. La banque centrale russe elle-même est bannie de toute transaction et ses avoirs en devises ce qui a provoqué l'effondrement du rouble. J'ai pu m'entretenir précédemment avec mes homologues des pays frontaliers de l'Ukraine et de la Russie : tous sont satisfaits de cet arsenal inédit de sanctions. En complément, l'Union s'est mobilisée pour soutenir l'Ukraine. Elle a activé la Facilité européenne pour la paix (FEP), ce nouvel instrument extrabudgétaire de réponse aux crises internationales, qui est dotée de 5 milliards d'euros

de mettre les règles de l'espace Schengen entre parenthèses pour ne pas entraver les ressortissants ukrainiens fuyant la guerre. En outre, le Conseil a déclenché le dispositif intégré de l'Union européenne pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise de crise (IPCR) afin de permettre une prise de décision rapide et coordonnée, comme lors de la crise migratoire de 2015, puis pour faire face à la pandémie. Les ministres se sont aussi entendus pour accorder la protection temporaire à l'ensemble des ressortissants ukrainiens qui ont trouvé refuge dans les États membres, sans préjuger de leur qualité de réfugiés. Au-delà de l'urgence, cette crise ébranle profondément l'Union, qu'il s'agisse de sa sécurité, de son équilibre, de son unité ou même de son identité. Tout d'abord, nous vivons un moment déterminant pour la sécurité de l'Union européenne. Si l'Ukraine tombe, nul ne sait où l'agresseur va s'arrêter. va s'arrêter. Le peuple ukrainien mène son combat pour toute l'Europe : en défendant sa liberté, il défend la nôtre. C'est pourquoi nous lui devons reconnaissance, admiration et soutien.

réfugiés. Selon l'ONU, à l'heure où nous parlons, 677 000 Ukrainiens ont déjà quitté leur pays. Plus de la moitié ont rejoint la Pologne, les autres la Hongrie, la Roumanie et la Slovaquie. L'Union européenne doit se préparer à une crise humanitaire d'une ampleur historique, touchant plus de 7 millions de personnes. Ce défi gigantesque frappe d'abord les pays limitrophes, lesquels nous ont déjà fait valoir les limites de leurs capacités d'accueil, malgré leur bonne volonté. Aujourd'hui, l'ensemble des États membres se disent prêts à accueillir les réfugiés ukrainiens, mais la question se posera rapidement de leur répartition entre les pays. La solidarité entre les États membres sera alors, une nouvelle fois, mise à rude épreuve. La crise ukrainienne aura aussi des répercussions économiques certaines : d'ores et déjà, elle renchérit encore davantage les prix de l'énergie.

a renoncé à mettre en service le nouveau gazoduc Nord Stream 2- ce dernier aurait privé l'Ukraine des ressources qu'elle tire du transit sur son sol du gaz russe exporté vers l'Union. Cette crise exige de penser la transition énergétique au prisme de l'autonomie stratégique. Elle annonce des hausses de prix accrues pour les Européens, si bien que la Commission européenne envisage de développer la « boîte à outils » qui, depuis l'automne dernier, permet aux États de répondre à la crise de l'énergie par des aides publiques et des abattements fiscaux. Se profilent aussi une flambée des prix des matières premières, y compris agricoles, des difficultés d'approvisionnement de certaines filières industrielles européennes en composants et métaux critiques, comme le titane ou le nickel, des ruptures dans les chaînes de production européennes en Russie, sans compter l'impact des représailles russes, qu'il faudra bien sûr assumer. L'Union européenne revoit d'ores et déjà à la baisse ses prévisions de croissance, de l'ordre de 0,3 % à 1 %, et l'inflation s'accentue encore après le record de ce mois de janvier. Un dernier défi défi ébranle l'Union : la demande officielle de l'Ukraine d'entrer sans délai dans l'Union européenne. La présidente de la Commission européenne a répondu hâtivement de façon positive, rejointe par plusieurs États membres d'Europe centrale. cette demande reflète la volonté majoritaire du peuple ukrainien ; mais nous parlons de décisions qui engagent durablement et qui, de ce fait, doivent être mûries. Ce n'est pas un hasard si la procédure d'adhésion est un processus au long cours il faut du temps pour rapprocher la législation du pays candidat du droit européen et remplir différents critères, comme la stabilité politique ou une économie de marché viable. C'est aussi pourquoi la décision même d'octroyer à un État le statut de pays candidat relève de l'unanimité des N'oublions pas que les trois pays baltes ont dû patienter près de neuf ans pour entrer dans l'Union et que quatre pays des Balkans occidentaux, officiellement candidats, sont bloqués depuis des années dans l'antichambre de l'Union européenne, sans compter les deux autres, qui ne sont encore que candidats potentiels. L'Ukraine, elle, est liée à l'Union européenne par un accord d'association signé en 2014 dans le cadre du partenariat oriental, qui concerne aussi la Moldavie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Géorgie et le Belarus. Lancé en 2009 par l'Union, ce partenariat propose des relations économiques et politiques plus étroites en échange de réformes, mais sans promesse d'adhésion. Je rappelle que la tragédie que traverse l'Ukraine depuis novembre 2013 a commencé par une manifestation pro-européenne, en réaction à la décision du président d'alors de ne pas signer l'accord d'association avec l'Union européenne, document paraphé dès mars 2012. C'est ce qui a conduit au changement de gouvernement et aux élections législatives d'octobre 2014, lesquelles ont porté au pouvoir des partis réformistes pro-européens. Cet accord d'association, qui prévoit un libre-échange complet, offre de nouveaux débouchés économiques tant à l'Union qu'à l'Ukraine. Il a permis à l'Union de conforter sa position de premier partenaire économique de l'Ukraine : en 2019, le volume des échanges bilatéraux s'élevait à 43,3 milliards d'euros et l'Union représentait plus de 40 % du total des échanges commerciaux de l'Ukraine. En outre, depuis 2014, l'Union européenne et ses institutions financières ont mobilisé plus de 15 milliards d'euros sous la forme de subventions et de prêts. nous devons miser sur cet outil- le partenariat oriental -, qui a fait la preuve de son efficacité et peut nous permettre de renforcer sans délai le soutien de l'Union à l'Ukraine. Parallèlement, la construction de l'Union européenne doit se poursuivre sans que nous soyons aveuglés par l'urgence : c'est un projet de long terme, qui doit rester au service de la promotion des valeurs européennes. Soyons actifs, mais prudents. La véritable urgence, c'est d'assurer la désescalade ; c'est de rétablir la paix sur le sol ukrainien. Ce sera l'honneur de l'Union européenne !

L'invasion dramatique de l'Ukraine par la Russie a rebattu en un instant toutes les cartes géopolitiques, changé nos références et bouleversé nos perspectives. Il nous faut maintenant dresser un constat lucide de la situation, en tirer les conséquences et déterminer enfin dans quelle voie il convient d'avancer. Le constat, c'est d'abord celui d'un véritable choc de valeurs. En effet, nous assistons à une mobilisation puissante, déterminée et rapide de l'ensemble des démocraties occidentales contre la guerre, contre cette guerre inutile et sale voulue par un homme seul. Très clairement, les gouvernements et, désormais, les opinions publiques de nos pays ont conscience qu'il s'agit d'une agression contre la démocratie et contre la liberté. Les Ukrainiens veulent vivre libres : Vladimir Poutine ne le supporte pas.

Même la Suisse décide de s'aligner sur l'ensemble des sanctions européennes. Le monde du sport, d'habitude réfractaire à toute idée de positionnement politique, exclut la Russie de toutes les compétitions. Face au dynamitage de l'architecture de sécurité conçue à la fin de la guerre froide, ceux qui, comme nous tous, ont cru à la possibilité et même à la nécessité de dialoguer avec la Russie de Vladimir Poutine doivent aujourd'hui se rendre à l'évidence

à lui interdire les choix de société qu'il entend faire. Les Ukrainiens ont choisi collectivement de vivre selon un modèle démocratique, et c'est leur droit. La conséquence de ce constat, c'est qu'en cinq jours, par cette folle action, Poutine a tiré l'OTAN de sa léthargie. Il a fait avancer la défense européenne de trente ou cinquante ans, en réveillant l'esprit de défense qui sommeillait dans le coeur des Européens. Aujourd'hui, il semble que le pouvoir russe soit surpris par la vigueur et l'unanimité des réactions occidentales. C'est bien là le coeur du problème. Les régimes autoritaires sont profondément convaincus que les démocraties sont faibles et incapables de faire face à la violence. C'est une profonde erreur, mais elle se paye au prix fort. Ce soir, près de 700 000 réfugiés sont sur les routes et des milliers de morts sont déjà à déplorer.

Alors que les Russes viennent de bombarder la tour de la télévision ukrainienne pour faire taire les médias, pour faire taire la voix de l'Ukraine libre, il faut que le peuple ukrainien le sache : nous continuerons d'entendre sa voix, d'entendre la voix dénonçant les crimes qu'il subit. Contrairement à nos démocraties, Poutine n'accorde que peu d'importance et de valeur à la vie humaine et aux libertés. Son bilan effroyable en Tchétchénie, dans les conflits gelés, avec ses milices ou contre ses opposants, en donne une sinistre illustration.

C'est un facteur de risque supplémentaire, ainsi qu'une preuve que le dessein de Vladimir Poutine dépasse largement la seule Ukraine. Poutine sera au moins parvenu à ce résultat : rendre à l'Europe son unité et sa détermination.

Cela changera-t-il la donne en Méditerranée ? Il est sans doute trop tôt pour le dire. Du moins le monde entier voit-il qu'un coup de force militaire est une option qui peut se révéler très coûteuse. C'est aussi cela, l'enjeu de cette crise l'affirmation par les pays occidentaux que le droit international existe et que nous pouvons le faire respecter si, ensemble, nous le voulons. Tirons immédiatement les conséquences de cette nouvelle donne

marquait une remontée salutaire de notre effort de défense. Mais le monde a changé plus vite que nous ne l'avions prévu et nous devons accélérer la réponse au sujet de nos points plus faibles. Ainsi, nous devons faire un énorme effort pour augmenter nos stocks de munitions, en particulier de munitions complexes. sur Kharkiv, des lance-roquettes russes tirent en une minute ce qu'un régiment français tire en un an à l'entraînement, nous devons bien sûr réagir tous ensemble. De même se pose la question de notre aviation de combat.

nous ne pouvons rester au niveau envisagé. Il en est de même pour les frégates de la marine. Dans les trois armées, il nous faut fournir les efforts nécessaires pour que nos forces gagnent en masse et en épaisseur. C'est indispensable pour faire face, le cas échéant, à des conflits de longue durée.

Mais ces chiffres considérables doivent surtout nous inciter à construire avec elle, comme avec tous nos voisins européens, cette Europe de la défense qui renforcera notre sécurité collective.

autre urgence : la protection des frontières de l'Union et de nos amis et alliés de l'Est- États baltes, Pologne, Moldavie, Géorgie et Roumanie. La France est présente auprès de ses alliés et

Il nous faudra donc faire des choix collectifs. L'exécutif qui sortira des élections du printemps prochain sera confronté à toutes ces questions, dont la première sera : comment aller plus loin que la loi de programmation militaire actuelle

de 2023. Sans doute faudra-t-il faire plus encore. C'est à ce prix que nos coopérations européennes élargies pourront être à la hauteur des menaces nouvelles qui émergent. Le drame affreux que vit l'Ukraine doit nous servir de leçon. Bien sûr, notre diplomatie doit être renforcée dans ses moyens et dans son statut pour prévenir et écarter de tels dangers. Dans les moments extrêmes comme celui que nous vivons,

car il faudra bien que, tôt ou tard, la diplomatie succède à la violence. Il faudra rebâtir une architecture de sécurité pour l'Europe et assurer le retour à une paix durable.

En soutenant l'Ukraine contre cette agression inqualifiable, nous agissons pour que cesse au plus vite ce martyre. Mais nous montrons aussi au reste du monde

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, ce débat au titre de l'article 50-1 de la Constitution fait honneur à notre pays. Il lui fait honneur, car il marque l'unité de la Haute Assemblée pour témoigner au peuple ukrainien et à ses courageux dirigeants l'amitié, la solidarité et le plein soutien du peuple français. Le 24 février dernier, la Russie a lancé une attaque illégale et massive contre l'Ukraine. Cela fait maintenant six jours que l'armée ukrainienne et le peuple ukrainien se battent avec courage et héroïsme contre l'agresseur.

malgré tous les efforts diplomatiques déployés, au premier rang desquels ceux du chef de l'État. Tout d'abord, je tiens à vous indiquer très rapidement ce que nous observons. Nos moyens de renseignement, notamment nos satellites, nous permettent d'avoir une appréciation souveraine de la situation, que nous communiquons bien sûr à nos alliés. Ce que l'on peut dire à cette heure, c'est que les Russes poursuivent leur offensive sur tous les fronts au sud, depuis la Crimée ; dans l'est, depuis le Donbass, en appui des forces séparatistes ; et au nord, où ils mènent une offensive importante. Kiev est encerclée et des frappes sont en cours. Les frappes des premiers jours ont principalement ciblé des équipements, des infrastructures militaires et stratégiques. Le but, pour la Russie, était de conquérir la supériorité aérienne. Mais aujourd'hui la situation est plus confuse et les informations sont difficiles à vérifier. Les forces russes maintiennent un blocus naval en mer Noire et en mer d'Azov. Face à cela, nous avons de bonnes raisons de penser que les forces armées ukrainiennes résistent bien. Elles livrent des combats acharnés et font mieux face à l'invasion que ce que les Russes avaient anticipé. Cette combativité est le reflet du courage de tout un peuple, qui s'est levé pour défendre son indépendance et ses valeurs, lesquelles sont aussi les nôtres. J'en viens maintenant à ce que nous faisons, aussi bien à titre national qu'avec nos partenaires et nos alliés. Nous agissons dans deux directions : tout d'abord, pour aider les Ukrainiens à se défendre ; ensuite, pour assurer notre posture de défense, afin que la Russie comprenne bien à quoi elle s'exposerait si elle s'en prenait à l'Alliance. Comme vous le savez, un engagement direct de nos forces ou de celles de nos alliés pour soutenir l'armée ukrainienne face à la Russie n'est pas une option. Il ferait de nous des cobelligérants de ce conflit. Or un pays comme la France ne peut recourir à la force que s'il est directement attaqué ou dans le cadre des alliances auxquelles il appartient. Pour autant, nous ne pouvons pas rester les bras croisés et laisser la résistance ukrainienne démunie face à un ennemi résolu à l'écraser, au mépris de toutes les règles du droit international. C'est pourquoi nous avons décidé de répondre à l'appel de l'Ukraine et de lui livrer des équipements de défense. Vous le comprendrez aisément, je ne puis en donner ici le détail.

C'est la première fois que la Facilité européenne de paix est utilisée depuis sa création, il y a un an, après des mois d'efforts auxquels la France a pris toute sa part. cette Facilité européenne de paix n'a pas surgi miraculeusement des tiroirs des bureaux bruxellois : c'est le résultat des efforts engagés sous l'impulsion du Président de la République dès le discours de la Sorbonne, en septembre 2017. C'est donc un pas historique pour l'Europe, qui a su agir vite et fort. À l'heure de la présidence française du Conseil de l'Union européenne (PFUE), nous sommes déterminés à aller encore plus loin pour donner à l'Europe de la défense tous les outils dont elle a besoin. Nous avons aussi décidé hier, avec l'ensemble des ministres de la défense européens, des moyens de coordonner nos aides bilatérales à l'Ukraine. L'état-major de l'Union européenne a été désigné pour répondre aux demandes ukrainiennes, qu'il s'agisse des équipements de protection, des armements ou des munitions. L'Union européenne va également pouvoir s'appuyer sur un logistique en Pologne. Comme vous le savez, la France est un contributeur majeur à la sécurité de ses alliés. Au lendemain de l'annexion illégale de la Crimée par la Russie en 2014, les chefs d'État et de gouvernement de l'Alliance atlantique s'étaient accordés pour le déploiement d'une présence avancée renforcée dans les États baltes et en Pologne. Il s'agissait de montrer à tout agresseur potentiel que le territoire des pays baltes et de la Pologne était bien couvert par la garantie de l'Alliance nous y avons pris toute notre part depuis le début et nous continuons de le faire. La situation créée par l'agression russe nous a conduits à décider le renforcement de ces dispositifs, sens d'une escalade, mais tout simplement pour défendre et rassurer nos alliés de l'Est. Le Président de la République a été très clair lors du Conseil européen, jeudi dernier, et lors du sommet de l'Alliance atlantique, le lendemain. Nous allons donc accélérer et renforcer le déploiement déjà prévu de nos avions de chasse dans les États baltes. Dès la mi-mars, quatre Mirage 2000, appuyés par une centaine d'aviateurs, seront déployés en Estonie. le 24 février, des patrouilles quotidiennes de deux Rafale et d'un avion ravitailleur s'envolent depuis la France pour réaliser des patrouilles dans les espaces aériens situés sur le flanc Est de l'Europe. Par ailleurs, nous renforcerons ponctuellement notre dispositif en Estonie, où une compagnie d'infanterie de montagne, composée de 200 militaires, sera déployée aux côtés de nos alliés danois et britanniques. nous avons accéléré le déploiement de moyens en Roumanie dans le cadre de l'OTAN, comme le Président de la République l'avait proposé dès le mois de janvier

Pour terminer, je souhaite partager avec vous quelques réflexions sur ce à quoi nous nous préparons. La crise que nous vivons a fait brutalement prendre conscience à l'opinion publique que la guerre n'était pas une réalité se résumant à des conflits asymétriques sur des théâtres éloignés. L'invasion de l'Ukraine et les menaces proférées par le président Poutine à notre égard montrent que notre sécurité se joue directement en Europe. Ce constat- vous le savez bien, ici, au Sénat -n'est pas nouveau pour le ministère des armées. Dès 2017, dans le cadre du travail stratégique engagé pour préparer la loi de programmation militaire, nous avions décrit le retour des stratégies de puissance et leurs conséquences.

qui nous a conduits à poser trois questions et, surtout, à commencer d'y répondre. Tout d'abord, quelle est notre crédibilité face à un agresseur puissant et déterminé ? C'est tout l'enjeu de la remontée en puissance de notre outil de défense. Après des décennies de sous-investissement, la dernière loi de programmation militaire a précisément inversé la tendance pour moderniser nos forces et pour sécuriser un modèle d'armée complet à l'horizon de 2030. Ensuite, quelle est notre capacité à agir en commun avec nos alliés et nos partenaires ? Soyons clairs, il y a peu d'hypothèses dans lesquelles la France serait engagée seule dans un conflit de haute intensité. Les mesures que j'ai évoquées, il y a un instant, montrent à quel point notre engagement au sein de l'Union européenne comme de l'Alliance atlantique est une composante essentielle de notre défense.

massives ou des tentatives qui viseraient à paralyser nos satellites, ce qui n'est pas une situation totalement inédite. Mesdames, messieurs les sénateurs, nous vivons, vous l'avez tous dit, un moment historique. historique pour l'Ukraine, qui lutte pour sa survie en tant que Nation et pour les valeurs que tous les Européens ont en partage. Il l'est aussi pour l'Europe, qui doit être à la hauteur. Soit l'Europe fait face, soit elle s'efface. Avec les mesures très fortes prises au cours de ces derniers jours,

1992, Kharkiv et Kiev aujourd'hui : l'Ukraine s'ajoute à la liste tragique des cauchemars européens.

ce sens, le 24 février 2022 restera dans l'Histoire, et au regard de l'Histoire, comme le jour d'une régression majeure dans la vie internationale et le droit international. Le jour où, en Europe, la Russie est revenue sur le primat du droit sur la force, alors même qu'elle est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies. Le jour où, en Europe, la Russie a voulu anéantir la souveraineté d'un État. Le jour où, en Europe, la Russie, en lançant une guerre contre 44 millions d'Ukrainiens, a affiché son mépris des droits humains les plus fondamentaux, comme le disait le président Cambon, les droits « à la vie, à la liberté, à la sûreté de sa personne », tous reconnus par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Le président Retailleau rappelait combien il était nécessaire de repenser le multilatéralisme pour le rendre plus efficace, en faisant preuve d'imagination. C'est

Il a refusé la voix de la diplomatie, il n'a pas tenu les engagements qu'il avait pris- le Premier ministre l'a rappelé -, il n'a pas honoré la signature de la Russie, il a menti : il porte donc seul l'entière responsabilité de sa décision d'engager cette guerre.

le seul gouvernement légitime de l'Ukraine est issu des urnes : c'est celui du président Zelensky. C'est lui et lui seul que nous reconnaissons et il n'est pas question d'adopter une autre position, ni aujourd'hui ni demain.

au profit des populations qui sont victimes du conflit. Un premier envoi de 33 tonnes de matériel est arrivé aux frontières de la Pologne, hier. Aujourd'hui, deux rotations aériennes ont permis d'acheminer 8 tonnes de matériel médical

sur l'activation du dispositif de protection temporaire, sur l'extension des visas pour les personnes qui sont présentes sur notre sol, et sur le travail que les préfets conduiront avec les collectivités locales pour recenser toutes les propositions en matière d'accueil et d'hébergement.

isolé la Russie, puisqu'elle a été le seul État à voter contre la résolution que nous avons portée avec 82 autres

Pour ce qui concerne les sanctions, je serai bref. M. le Premier ministre l'a dit dans son intervention liminaire, l'Union européenne a pris trois paquets de sanctions. Un quatrième paquet a été décidé le 28 février au soir pour intégrer la Biélorussie, en tout cas des acteurs biélorusses, dans le champ des sanctions.

Nous devons, après chaque décision du Conseil en matière de sanctions, attendre la mise en place du règlement y afférent. Nous y travaillons activement, afin de préciser le champ des actifs et des avoirs que nous voulons geler ou saisir, la nature exacte des marchandises interdites ou des trafics interdits, et les modalités d'intervention. Je peux vous assurer de la détermination et de la mobilisation des services de l'État pour procéder à ces gels et à ces sanctions dans le cadre des règlements déjà publiés. Des navires ont d'ores et déjà été arraisonnés, et font l'objet d'un gel. Des avoirs sont en cours d'identification, également en vue d'un gel. Nous avons appris avec beaucoup de satisfaction l'accord de la Suisse pour transposer dans son droit interne la totalité des règlements des sanctions prises par l'Union européenne, mais aussi l'accord de la Principauté de Monaco.

l'a dit -, par une assistance macroéconomique de 1,2 milliard d'euros accordés par l'Union européenne, ainsi que par une aide directe de la France à hauteur de 300 millions d'euros. Comme le Président de la République s'y est engagé, nous veillons évidemment à la traçabilité de ces aides. Nous veillerons aussi à ce qu'elles soient accordées au gouvernement ukrainien légitime ; cela implique évidemment de suivre l'évolution de la situation en Ukraine, ce que nous faisons. J'en Ukraine, ce que nous faisons. J'en viens à la question des conséquences économiques pour la France. L'économie française n'est pas l'économie la plus exposée aux difficultés liées aux échanges avec la Russie.

celui de la chimie, de la parfumerie et de la cosmétique, pour 21 % ; celui de la pharmacie, pour 12 % ; celui des machines industrielles et agricoles, pour 10 %. Nous portons une attention particulière, qui a été rappelée ici même et à l'Assemblée nationale, au secteur de l'agroalimentaire,

Quel sera l'impact sur les finances publiques de ces différentes mesures ? Il est évidemment trop tôt pour le savoir, et ce pour deux raisons. Premièrement, nous ne savons pas mesurer, à ce stade,

concerné par l'augmentation du prix du gaz, puisque certaines centrales thermiques fonctionnent grâce au gaz. Surtout, les mécanismes de régulation du marché européen de l'électricité indexent largement le prix de l'électricité sur le prix du gaz. Nous répondrons à cette situation, M. le Premier ministre l'a dit, en prolongeant autant que nécessaire le bouclier tarifaire concernant le gaz et l'électricité, que nous avions mis en place pour faire face à une autre crise de l'énergie. Il peut s'avérer utile pour protéger les ménages. Nous aurons également à traiter la question des entreprises,